proposition de résolution invitant à favoriser la restauration de la sécurité en Haïti afin de créer les conditions nécessaires à la mise en place d’un processus politique de sortie de crise présentée, en application de l’article 34 1 de la Constitution, par Mme Hélène Conway Mouret

je me réjouis de porter enfin devant vous cette proposition de résolution invitant à favoriser la restauration de la sécurité en Haïti, afin de créer les conditions nécessaires à la mise en place d’un processus politique de sortie de crise. Un long intitulé, pour une belle ambition. Nous avions travaillé à la rédaction de ce texte il y a plus de dix huit mois, déjà convaincus de l’urgence de la situation et de l’absolue nécessité de mobiliser davantage la communauté internationale pour venir en aide à ce pays avec lequel nous avons noué, au fil de l’histoire, une relation unique. Comment qualifier l’urgence, lorsqu’elle se prolonge si longtemps, que les cris et les pleurs du peuple haïtien ne transpercent plus le mur des médias, et que nous semblons comme accoutumés au désespoir ?

Depuis des mois, le groupe d’amitié France Caraïbes du Sénat, que j’ai l’honneur de présider, a mené des auditions, accueilli des conférences, travaillé avec le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, avec l’ambassadeur de France à Port au Prince et l’ambassadeur d’Haïti à Paris, dont je salue la présence dans nos tribunes pour suivre nos discussions. J’ai échangé avec le président du conseil présidentiel de transition haïtien Leslie Voltaire, lors de sa venue à Paris le 29 janvier dernier. Nous avons aussi rencontré la délégation haïtienne à l’occasion du dernier sommet de la Caricom, la Communauté caribéenne, en février 2025, dans le but d’alimenter notre réflexion et de déterminer les axes d’action prioritaires pour accompagner Haïti à la mesure de ses besoins actuels et des exigences de l’histoire qui nous unit.

D’une même voix, nous demandons un engagement fort de notre pays et de la communauté internationale en faveur de la restauration de la sécurité en Haïti, condition indispensable à toute sortie de crise politique durable dans ce pays frère, meurtri et épuisé, mais digne et résilient. Nous le devons à ce peuple qui, peut être plus que tout autre, a fait siens les idéaux universels portés par les Lumières. La quête de liberté, le respect de la dignité humaine, la lutte contre l’oppression sont autant de valeurs que nous avons en partage et qui nous obligent mutuellement, mutuellement, créant entre nos deux pays un lien indéfectible qui traverse les siècles. L’humanité du peuple haïtien, blessé et malmené par tant de violence, nous invite à réagir. N’oublions pas que la France est aussi un pays caribéen, et que nos territoires d’outre mer sont aux premières loges du désolant spectacle de l’effondrement d’Haïti. Si nous ne réagissons pas fortement, nous savons que nous nous mettons en danger pour l’avenir. La violence ne pourra pas éternellement être circonscrite à ce qu’on appelait la perle des Antilles, que nous souhaiterions voir retrouver tout son lustre. lustre. Je rappelle quelques chiffres, derrière lesquels se cachent autant de vies humaines, de destins brisés. Les gangs armés ont pris le contrôle de pans entiers du territoire, notamment à Port au Prince. Ainsi, plus de 80 % de la capitale serait désormais sous leur domination. Ces groupes se livrent à des affrontements sanglants ; ils contrôlent l’accès aux routes, aux ports, aux quartiers. Ils ont même fermé l’aéroport pour un temps et commettent enlèvements, viols collectifs, assassinats ciblés et extorsions. Les violences ont fait des milliers de morts pour la seule année 2024, au moins 5 601 personnes ont été tuées, 2 212 blessées et 1 494 kidnappées. Ce sont des chiffres de temps de guerre. Et pourtant, ce conflit ne dit pas son nom. Parce qu’il n’y a pas de limite à l’horreur, les violences sexuelles sont désormais utilisées comme des armes. En recourant aux viols collectifs, c’est la soumission des communautés qui est recherchée, c’est l’espoir d’une reconstruction qui est anéanti. Dans ce pays, qui est aussi victime d’une série noire de catastrophes naturelles – rappelons les 280 000 morts ayant suivi le séisme de 2010, ainsi que les destructions et pertes humaines causées par les ouragans qui s’abattent régulièrement sur l’île –, la violence vient aggraver la crise humanitaire. Là aussi, les chiffrent donnent le tournis : on compte un million de déplacés internes, soit 9 % de la population ; près de la moitié de la population est en insécurité alimentaire ; la recrudescence du choléra fait des dizaines de victimes, en particulier chez les enfants de moins de 5 ans ; 80 000 personnes sont infectées par le VIH, que seuls 28 % des établissements d’hospitalisation sont pleinement opérationnels. Le défi humanitaire est immense, et la France participe à une coalition des volontaires, notamment au travers des 16 millions d’euros d’aide humanitaire versés en 2024. Cependant le désengagement américain rebat les cartes de la solidarité internationale. Il nous oblige à revoir et à accentuer notre effort aux endroits où l’urgence est la plus absolue. Haïti fait partie des priorités.

Sans avancée décisive dans ce domaine, c’est tout le fonctionnement démocratique, économique et social du pays qui se trouve empêché. Une première étape a été franchie avec la résolution du 2 du 2 octobre 2023 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui autorise la constitution et le déploiement d’une mission multinationale d’appui à la sécurité. Le Kenya a pris la tête de cette force, et un an et demi plus tard, un millier de policiers étrangers sont présents sur le terrain : 750 policiers kenyans, 150 militaires guatémaltèques, 75 militaires salvadoriens et 25 policiers de Jamaïque, des Bahamas et du Bélize. Mais ce déploiement est trop lent, les forces policières sont sous équipées et elles ne parviennent pas à enrayer les violences, malgré le courage exceptionnel de leurs hommes, que je tiens ici à saluer. L’un des obstacles majeurs est le financement de la mission, qui repose aujourd’hui uniquement sur les contributions volontaires des États. Ainsi, sur les 110 millions de dollars versés par les États membres depuis la création de la mission, le Canada apparaît comme le premier contributeur, à hauteur de 63 millions de dollars, suivi par les États Unis, 15 millions de dollars. La part de la France s’est élevée à 8 millions d’euros en 2024. À cela s’ajoutent les autres aides, versées directement par les États sans passer par le fonds onusien. Ainsi, les États Unis de l’administration de Joe Biden avaient engagé plus de 300 millions de dollars en fonds et en équipements destinés à la mission multinationale, dont des dizaines de véhicules blindés. La France a, elle, consacré 2 millions d’euros en 2024 au soutien à la police nationale haïtienne et aux forces armées d’Haïti, car le renforcement des capacités locales est une condition indispensable à l’émergence de solutions pérennes. Au regard de l’ampleur de la tâche à accomplir, de la poussée des gangs depuis la fin de l’année 2024 et de l’incertitude qui pèse sur la pérennité des contributions américaines, la communauté internationale n’a d’autre option que d’accentuer son effort. S’il n’existe pas de majorité au sein du Conseil de sécurité des Nations unies pour avancer vers une véritable opération de maintien de la paix, comme le demande le gouvernement de transition haïtien, il nous faut réfléchir à des solutions de remplacement qui permettront de répondre au besoin de sécurisation des financements. La proposition du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies d’avancer vers un format hybride en créant un bureau de soutien de l’ONU permettrait de financer directement, sur budget onusien, toute la logistique liée à la mission internationale, notamment pour le logement, la nourriture, le transport et les communications. Pouvez vous nous indiquer, monsieur le ministre, si la France appuiera l’adoption rapide de la proposition du secrétaire général de l’ONU ? Au delà de cette réflexion de fond, quel sera le montant de la contribution française à la mission multinationale en 2025 ? chers collègues, nous avons aujourd’hui un devoir de fraternité, une responsabilité partagée. Car Haïti, terre de fierté et de douleur, a plus que jamais besoin d’un partenaire ambitieux dans sa vision et constant dans son engagement.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Sénat lance cet après midi une nouvelle alerte une nouvelle alerte face au drame humain, sécuritaire, politique, environnemental, économique et social qui se joue dans le pays le plus peuplé des Caraïbes ; une nouvelle alerte qui traduit aussi notre capacité collective à adopter, au delà de nos appartenances politiques des positionnements qui rassemblent l’ensemble des sensibilités républicaines représentées dans cet hémicycle. Je veux, à cet égard, saluer l’initiative défendue par ma collègue Hélène Conway Mouret, auteure de cette proposition de résolution, s’inscrit dans le prolongement de son engagement de longue date en faveur de la restauration de la sécurité en Haïti. Haïti, un pays avec lequel la France partage des liens intimes, tissés au fil d’une histoire commune, une histoire aux pages teintées de lignes sombres, trop longtemps tue ; des liens étroits, cultivés à travers une langue partagée et à travers une relation récemment restaurée.

marqué par les séquelles de la colonisation et de l’esclavage, est l’une des premières voix de la liberté, de l’indépendance et de l’abolition. Haïti est un État avec lequel la France a depuis plusieurs années engagé une coopération étroite, une coopération étroite, que nous devons à présent renforcer, à la fois en termes d’appui sécuritaire et d’aide humanitaire, tant la situation sur place est accablante et le contexte international propice à l’enlisement du pays dans la pluralité des crises auxquelles il est confronté. Il y a une semaine, à Mirebalais, commune située au nord est de la capitale de Port au Prince, les gangs armés, qui contrôlent deux des dix départements du pays, soit 50 % de la population, confirmaient qu’ils n’ont d’autre stratégie que de propager le chaos et le déchaînement de la violence. Le tableau est glaçant : un assaut contre un établissement pénitentiaire, 529 détenus évadés, des policiers en sous effectif fuyant le commissariat, des morts, des blessés parmi la population locale, contrainte de se réfugier dans les communes voisines, des autorités débordées et des bandes criminelles sur le point de prendre le contrôle de nouveaux territoires et de s’emparer d’infrastructures clés. Ce nouvel affrontement confirme que l’île est au centre d’un cataclysme sécuritaire, comme en témoignent les 5 601 personnes tuées en 2024. L’auteure du texte l’a rappelé Au nom du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, je veux à cet instant avoir une pensée pour la population haïtienne, touchée par l’assassinat de son président Jovenel Moïse en juillet 2021, puis par une crise ravivée par la démission en mars 2024 du Premier ministre Ariel Henry une population victime d’assassinats, de viols collectifs, d’enlèvements et de pillage ; une population marquée à jamais par les terribles séismes de janvier 2010 et d’août 2021.

déjà le cas durant trois semaines en novembre 2024, en raison des affrontements de rue qui ont lieu à quelques encablures de nos installations. Face à l’ampleur de la crise, la tenue de ce débat témoigne d’une véritable prise de conscience. La proposition de résolution soumise à notre examen confirme combien il est urgent de venir en aide à la population haïtienne et de restaurer la sécurité dans le pays,

L’accord politique pour une transition pacifique et ordonnée, conclu le 3 avril 2024, fait d’ailleurs de la sécurité une priorité. Les chiffres parlent d’eux mêmes : avec un membre d’une force civile ou militaire pour mille habitants, les effectifs sont structurellement insuffisants, ce qui crée un rapport de force favorable aux gangs. Dans ce contexte, nous nous associons pleinement à l’appel lancé par notre collègue Hélène Conway Mouret visant à conforter le soutien de la France au déploiement de la mission multinationale d’appui à la sécurité de la police nationale haïtienne, mise en place en 2023 sous l’égide des Nations unies. Cette mission compte à ce jour un millier de membres de forces de l’ordre. La France a été au rendez vous de l’appui à la sécurité. Elle a mobilisé au total dix millions d’euros l’an dernier,

chers collègues, ce texte est aussi un appel au sursaut humanitaire, un appel à agir plus vite et plus fort en faveur du million de femmes, d’hommes, mais aussi de nouveau nés et d’enfants déplacés du fait de la violence des gangs

Face à la détérioration des conditions de vie de la population haïtienne, nous demandons une amplification du soutien de la France en termes d’aide humanitaire et alimentaire. En effet, 5,6 millions de personnes, soit près de la moitié de la population, se trouvent actuellement en situation d’insécurité alimentaire. Nous alertons également sur le risque pesant sur les personnes les plus vulnérables, susceptibles d’être recrutées demain par les gangs dont elles sont aujourd’hui les victimes. La promesse d’une vie meilleure au sein de ces bandes criminelles conduira mécaniquement à une spirale incoercible de violences. Là aussi, il est urgent d’agir, particulièrement au sein des camps de déplacés, qui pourraient bientôt être privés d’eau, de nourriture et de soins. la France a été au rendez vous de l’aide humanitaire, en mobilisant 16 millions d’euros et en finançant la construction de cantines scolaires dans neuf départements sur les dix que compte le pays. Cela représente 80 000 repas par jour, il faut le souligner. De solidarité, il a également été question l’an passé avec la mobilisation de 2 millions d’euros pour aider les sites accueillant les personnes déplacées et de 2 millions d’euros supplémentaires pour soutenir les Haïtiens renvoyés de la République dominicaine. Depuis octobre 2024, ils seraient 200 000 à avoir été confrontés à cette situation. Ce chiffre est préoccupant à l’heure où les États Unis multiplient eux aussi les procédures de renvoi. En matière d’aide humanitaire, nous devons à tout le moins poursuivre nos efforts et maintenir les crédits alors que les besoins financiers sont estimés à 908 millions de dollars en 2025, soit une augmentation de 35 % par rapport à 2024.

Pour ces raisons, et eu égard aux liens étroits tissés avec Haïti, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera naturellement cette proposition de résolution. Monsieur le ministre, je saisis l’occasion qui m’est les alertes que nous avons déjà lancées concernant les conséquences de la réduction des crédits consacrés à l’aide publique au développement. Si celle ci ne représente que 1 % du budget total de l’État, elle supporte à elle seule 10 % des coupes budgétaires en 2025, après une première réduction en 2024. Défendre l’aide publique au développement, c’est choisir l’investissement de long terme, c’est avoir la conviction que la prospérité et la stabilité des nations sont indissociablement liées, c’est agir concrètement et résolument en faveur des programmes vitaux pour la santé, pour l’éducation, pour l’assainissement, pour l’agriculture et pour le soutien aux droits des femmes.

Mouret, auteure de cette proposition de résolution, ainsi que par ses collègues du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Voilà maintenant un peu plus d’un an que le Premier ministre Ariel Henry a démissionné de sa fonction de chef de l’État haïtien par intérim, après avoir passé deux ans

désormais que la loi du plus fort. Les gangs s’y disputent le territoire en raison de la profusion d’armes à feu et leurs affrontements font de nombreuses victimes, tant au sein des bandes armées que parmi les civils.

Certaines sources font même état de traite d’enfants. La communauté internationale ne peut laisser faire cela. Ces drames n’épargnent aucun Haïtien. Durant le seul mois de mars, plus de 60 000 personnes ont été déplacées. Les forces de l’ordre locales, quant à elles, dépassées et démoralisées, basculent parfois du côté des gangs. Ainsi, Jimmy Chérizier, tristement célèbre, est passé de policier à chef de gang ; il a participé à des massacres, ainsi qu’à des attaques de prisons ayant conduit à l’évasion de près de 4 000 prisonniers. Face à cette situation, de nombreux Haïtiens fuient vers l’État voisin de Saint Domingue. Cette dynamique migratoire engendre des tensions croissantes avec la République dominicaine, où des manifestations hostiles aux migrants haïtiens se sont Haïti est devenu un enfer à ciel ouvert, livré aux mains de bandes armées. Ce chaos intervient après plusieurs catastrophes naturelles, tremblements de terre,

Alors que la situation est loin d’être sous contrôle, les États Unis, deuxième bailleur de cette mission, ont récemment annoncé la suspension de leur financement, infligeant un coup dur à une opération déjà fragile. Nos collègues soumettent aujourd’hui de résolution afin que cette tragédie ne tombe pas dans l’oubli et que des moyens soient mis en œuvre pour remédier à la situation. Tous les présidents de groupe de notre assemblée ont cosigné cette proposition, témoignage témoignage de notre unanimité sur ce sujet, dont le volet humain est fondamental. Il est souvent dit que la sécurité est la première des libertés ; Haïti en offre une

même devra sans doute être réexaminé après le gel du financement américain. Parallèlement aux efforts de maintien de l’ordre, la communauté internationale devra renforcer le soutien logistique, médical et humanitaire, restaurer la sécurité ne suffira pas. Il faudra également aider Haïti à reconstruire un tissu social, économique et institutionnel. cours de la reconstruction, il faudra veiller à créer les conditions d’une paix durable et à soutenir un renouveau politique fondé sur des processus démocratiques robustes. L’urgence aujourd’hui est au retour à l’ordre. Des moyens à la hauteur de la catastrophe doivent être engagés si nous entendons l’enrayer.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, oui à la fraternité internationale ! Évoquer Haïti, c’est avant tout témoigner d’un attachement jamais démenti à ce pays, où j’ai eu la chance de me rendre à l’occasion de huit missions entre 2009 et 2018, notamment quelques semaines avant, puis quelques semaines après, le séisme du 12 janvier 2010.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette proposition de résolution a pour ambition de donner une impulsion politique en faveur d’une intervention internationale et d’un soutien accru à Haïti, afin de rétablir la sécurité face aux violences et aux actes de barbarie commis envers la population civile par les gangs. Cette volonté, portée par notre diplomatie parlementaire, apparaît essentielle au regard de la situation chaotique dans laquelle Haïti des Caraïbes traverse l’une des pires crises de son histoire, marquée par une instabilité politique persistante, par une insécurité grandissante et par une catastrophe humanitaire alarmante. alarmante. Déjà fragilisé par des décennies de troubles politiques et de catastrophes naturelles, il fait désormais face à une détérioration sans précédent de ses conditions de vie. Les gangs armés contrôlent de vastes zones, notamment 80 % de la capitale, Port au Prince, où les enlèvements, les violences, les viols et les affrontements sont devenus monnaie courante. La population vit dans la peur constante et les forces de l’ordre, insuffisamment équipées et parfois corrompues, ne parviennent pas à rétablir l’ordre. La situation humanitaire est tout aussi dramatique. La pauvreté touche plus de 60 % de la population, et l’accès aux biens et aux services essentiels tels que l’eau potable, l’éducation et les soins de santé restent très limités. L’insécurité alimentaire atteint des niveaux critiques, près de la moitié des Haïtiens vivant en situation de sous alimentation.

le paiement d’une indemnité massive de 150 millions de francs or en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette somme exorbitante, équivalant à environ 21 milliards de dollars actuels, représentait à l’époque une indemnisation des colons pour la perte de leur outil de travail, autrement dit les esclaves.

d’Haïti. Ce lourd héritage nous oblige aujourd’hui à ne pas rester indifférents au sort d’Haïti, pays plongé dans une crise sans précédent dont il ne pourra sortir sans la solidarité internationale, notamment

Cette crise a en effet des répercussions majeures, en particulier en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Ces territoires partagent des liens historiques et culturels forts avec Haïti

Les préfectures des Antilles doivent gérer un nombre croissant de demandes d’asile, alors même que leurs services administratifs sont déjà saturés. Les centres d’hébergement d’urgence se trouvent souvent débordés les municipalités doivent faire face à la hausse des besoins en logement, en éducation et en soins pour ces nouveaux arrivants. Les systèmes de santé en Guadeloupe et en Martinique sont pourtant déjà fragilisés par des pénuries de personnel et des difficultés budgétaires les écoles locales, en particulier dans les quartiers où s’installent majoritairement les Haïtiens, sont saturées et doivent faire face à des défis linguistiques et pédagogiques, certains enfants ne maîtrisant pas suffisamment le français ou nécessitant une remise à niveau scolaire.

Pour le peuple haïtien, nous devons agir afin d’aider au rétablissement de la sécurité et de faciliter une transition démocratique.

Haïti est un pays brisé. Pays le plus pauvre des Amériques, il se trouve confronté, depuis des décennies, à une crise politique, économique, sociale et sécuritaire sans précédent, à laquelle viennent s’ajouter séismes, ouragans et épidémies. Ainsi, l’histoire récente d’Haïti est le récit d’une longue descente aux enfers.

Si l’on ajoute à cela l’occupation du pays par les États Unis au début du XX siècle, la corruption successive de ses dirigeants et les catastrophes naturelles, l’on comprend mieux pourquoi Haïti, perle des Antilles, figure désormais parmi les pays les plus pauvres du monde.

Le pays est plongé dans une profonde instabilité politique depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse en 2021, événement ayant accéléré la dégradation sécuritaire. La démission forcée du Premier ministre Ariel Henry l’année dernière n’a pas permis d’enrayer ce chaos politique et la spirale de la violence.

Les chiffres sont alarmants : on recense plus d’un million de déplacés internes et, selon les ONG présentes sur place, la moitié de la population souffre d’insécurité alimentaire. Autrement dit, Haïti est plongé dans une véritable crise humanitaire.

Pour nos compatriotes comme pour les Haïtiens, mais également pour l’ensemble des pays de la région, à commencer par la République dominicaine voisine, la restauration de la sécurité dans le pays constitue donc un enjeu vital. Tel est précisément l’objet de la proposition de résolution que nous examinons aujourd’hui ; je remercie notre collègue socialiste de l’avoir présentée. Sortir Haïti de la crise dans laquelle le pays est plongé nécessitera un effort international considérable. Un premier pas a certes été engagé avec la mission menée par le Kenya, mais celle ci reste insuffisante, pour ne pas dire désormais de passer à la vitesse supérieure en renforçant la police nationale haïtienne et en organisant un retour durable à la paix. Un embargo sur les armes ainsi qu’une lutte efficace contre leur trafic doivent être instaurés immédiatement, car Haïti n’en produit pas. Après cette réponse sécuritaire,

À l’heure où les États Unis se replient sur eux mêmes, il est essentiel que la communauté internationale utilise tous les moyens à sa disposition pour accompagner Haïti et l’aider à sortir de l’engrenage de la violence. La France, de par l’histoire qui la lie à ce pays, doit être motrice dans ce déploiement. Le groupe du RDSE votera évidemment cette proposition de résolution.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues,

touchant à la sécurité, à l’économie, à la politique, mais aussi, bien sûr, à l’humanitaire. Le pays, déjà éprouvé par des catastrophes naturelles dévastatrices telles que les séismes de 2010 et de 2021, peine à se relever.

Entre janvier et septembre 2024, au moins 3 600 personnes ont été tuées et 750 000 autres contraintes de fuir leur domicile.

La situation humanitaire est également désastreuse. Plus de la moitié de la population, soit 5,5 millions de personnes, souffre d’insécurité alimentaire aiguë ; 2 millions de personnes se trouvent en situation d’urgence alimentaire et près de 6 000 vivent dans des conditions de famine. La malnutrition, répandue notamment chez les enfants, emporte des conséquences dévastatrices sur leur développement et leur avenir.

de 70 %. Sur le plan économique, Haïti fait face à des défis immenses. Selon la Banque mondiale, plus de 64 % de sa population vit avec moins de 3,65 3,65 dollars par jour. La crise sécuritaire et l’instabilité politique rendent difficile l’accès aux ressources essentielles, en premier lieu alimentaires, pour une grande partie de la population. Le processus politique demeure fragile et les institutions publiques sont en ruines. L’instabilité politique s’est aggravée depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021, plongeant la nation dans un vide institutionnel préoccupant. La dernière élection présidentielle et les dernières élections législatives remontent à 2016, et le Parlement haïtien n’est plus opérationnel depuis janvier 2020. Les tensions entre le Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre ont conduit à des changements fréquents dans le gouvernement d’Haïti, compliquant encore plus la situation politique. La corruption et l’impunité sont omniprésentes, ce qui complique encore davantage la résolution de la crise. Les efforts de la police nationale haïtienne et de la mission multinationale d’appui à la sécurité mandatée par le Conseil de sécurité des Nations unies n’ont pas réussi à enrayer la violence. L’État perd inexorablement du terrain face aux gangs, qui étendent leur contrôle et imposent leur propre loi dans de nombreuses zones. La communauté internationale a un rôle crucial à jouer pour aider Haïti à sortir de cette crise. Tel est l’objet de la proposition de résolution transpartisane que nous examinons aujourd’hui. Il est en effet impératif d’accélérer le déploiement de la MMAS et de s’assurer que des mécanismes de conformité aux droits de l’homme sont pleinement en place. Ce déploiement est d’une impérieuse nécessité au regard de la situation humanitaire du pays et du poids des gangs. Il nous faut en effet accentuer la coopération policière entre la France et Haïti, notamment en faveur de la formation des policiers, mais aussi pour l’acheminement d’armes adaptées à la lutte contre les gangs. L’accord signé à Kingston il y a un peu plus d’un an, le 11 mars 2024, est un bon début.

La proposition de résolution appelle enfin à mener une action déterminée pour assurer un acheminement rapide et sécurisé de l’aide humanitaire en Haïti.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la situation en Haïti est dramatique, nous en convenons tous. Faute de moyens suffisants et d’un appareil institutionnel stable, l’État haïtien peine à assurer la sécurité de sa population. Les gangs armés, profitant du vide laissé par des institutions affaiblies, exercent une emprise très inquiétante sur de larges pans du territoire et sur une part toujours croissante de la société. Face à cette détérioration, le Gouvernement haïtien a sollicité en octobre 2022 l’appui d’une force multinationale, une initiative qui a été ensuite validée par le Conseil de sécurité des Nations unies. Une majorité des membres de notre groupe soutient le principe de ce déploiement, guidée par la conviction que chaque citoyen a droit à la sécurité et à la dignité. Toutefois, ce soutien ne doit pas nous dispenser d’un examen lucide et rigoureux du contexte. L’approche exclusivement sécuritaire qui s’exprime dans ce texte, de même que dans les documents annexes transmis aux membres du groupe d’amitié France Caraïbes, risque de réduire une crise profondément politique à une seule urgence humanitaire. L’histoire récente d’Haïti montre que les interventions armées étrangères, quoiqu’elles soient souvent motivées par de bonnes intentions, ont rarement permis de stabiliser durablement le pays. Plus d’une dizaine de missions se sont succédé en trente ans, sans parvenir à enrayer la spirale de l’instabilité. Leur échec tient souvent au caractère partiel de l’analyse faite des causes de la crise haïtienne. Il est essentiel de le souligner, l’insécurité est non pas une cause, La crise actuelle est le fruit d’un enchevêtrement de facteurs : effondrement institutionnel, corruption systémique, inégalités sociales criantes, absence de perspectives économiques et persistance d’une élite politique et économique exerçant un contrôle informel sur les rouages de l’État. Plusieurs rapports, dont certains émanent des Nations unies, mettent d’ailleurs en lumière les liens très étroits entre certains groupes armés et des figures influentes de cette élite. Dans ce contexte, une force internationale agissant sans véritable feuille de route politique ni coordination avec des acteurs légitimes risque de renforcer un déjà largement rejeté par la population. En effet, le gouvernement en place depuis depuis juillet 2021, non élu, ne bénéficie d’aucune légitimité démocratique et apparaît de plus en plus comme un exécutif soutenu seulement par l’extérieur. Le risque est grand qu’une telle mission, au lieu de renforcer les institutions, ne fasse qu’affermir une police décriée pour sa corruption et ses connivences supposées avec les gangs. L’expérience passée, notamment l’épidémie de choléra introduite par des Casques bleus et les cas documentés d’abus commis par ces mêmes troupes, appelle à une vigilance extrême, d’autant que les victimes de ces précédentes missions attendent toujours justice et réparation. La seule issue durable à la crise haïtienne passe par un processus politique inclusif et souverain. À cet égard, l’accord de Montana, élaboré par un large éventail d’organisations de la société civile haïtienne – syndicats, églises, associations de défense des droits humains, mouvements féministes – constitue une initiative sérieuse. Il propose une transition de rupture avec les pratiques actuelles, en vue d’élections libres et crédibles, et le rétablissement des trois pouvoirs de l’État. Enfin, il est urgent d’ouvrir un débat international sur la dette d’Haïti, à commencer par la dette dite de l’indépendance, imposée par la France au XIX siècle, qui a lourdement entravé le développement du pays. Toute stratégie d’aide internationale devrait intégrer l’annulation complète des dettes actuelles, mais aussi la reconnaissance de cette dette historique. En conclusion, nous ne pouvons nous contenter d’une réponse armée. Il faut une vision globale, respectueuse de la souveraineté du peuple haïtien et construite en partenariat avec les forces vives du pays. La sécurité, certes, mais jamais au détriment de la démocratie ! La parole

en matière socio économique : Haïti est le pays le plus pauvre des Amériques depuis des décennies, et 36 % de la population survivent avec moins de deux dollars par jour. Le pays est régulièrement frappé par des catastrophes naturelles, avec de très forts séismes, en 2010 et en 2021, des ouragans et des inondations. À chaque catastrophe, les morts se comptent par milliers et les services publics se retrouvent en lambeaux. La santé des Haïtiens s’en trouve très dégradée : la mortalité infantile et maternelle reste élevée, la faim est omniprésente et le choléra fait des ravages. Face à une telle crise humanitaire, la vie politique haïtienne connaît un chaos total. Depuis 2020, le pouvoir législatif a cessé de fonctionner, avec la fin du mandat de l’ensemble des députés, puis des sénateurs. L’année suivante, le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné, dans un contexte de guerre des gangs, de trafic de drogue et de corruption généralisée. Plusieurs millions de dollars étaient ainsi cachés dans la chambre du président Moïse. Depuis deux ans, il n’y a plus aucun élu en fonctions en Haïti ; la légitimité du Premier ministre par intérim, Ariel Henry, nommé quarante huit heures avant ce meurtre, est extrêmement faible. L’État haïtien est donc en déliquescence totale. Mais la nature a horreur du vide. Sans État, ce sont les mafias qui prennent le relais, assurant une sécurité toute relative en contrepartie d’un racket de la population. De nombreux groupes armés se disputent le territoire et s’affrontent pour le contrôle du trafic de drogue vers les États Unis. La violence est endémique : l’an dernier, plus de 5 600 personnes ont été tuées, plus de 2 200 blessées et près de 1 500 kidnappées. Port au Prince, la capitale, détient ainsi le macabre record de la ville la plus violente au monde. Un million d’Haïtiens ont dû fuir leur logement face à ce climat de terreur.

qui a donné naissance à la mission multinationale d’appui à la sécurité, est un premier pas positif. Comme souvent dans l’histoire d’Haïti, la France et les États Unis ont été les plus actifs dans ce processus. Les États Unis apportent notamment à la MMAS un soutien financier, logistique, de renseignement, de personnel et de matériel militaire. Toutefois, l’histoire des relations d’Haïti avec la France et les États Unis est si tragique que ces deux nations ont perdu toute légitimité pour prétendre résoudre les problèmes de l’ancienne Saint Domingue. Longtemps sous domination française, la perle des Antilles s’est libérée du joug de l’esclavage à partir de 1791, puis est devenue indépendante en 1804. Cette libération, portée par Toussaint Louverture et les Jacobins noirs, a envoyé un message d’espoir au reste du monde colonisé et nous a rappelé que la Révolution française n’est pas complète si elle ne s’applique pas aussi aux esclaves et aux colonies. Malheureusement, la France monarchiste de Charles X obligea ensuite les esclaves à rembourser leurs anciens maîtres, en menaçant Port au Prince de la flotte royale. Cet épisode honteux de l’histoire française, dont nous commémorerons dans quelques jours le bicentenaire, est totalement oublié chez nous. Il ne l’est pas en Haïti, qui a consacré 80 % de son budget au remboursement de cette dette illégitime pendant cent vingt deux ans. Depuis lors, le soutien de la France et des États Unis à la dynastie des Duvalier, de sanguinaires dictateurs qui ont ruiné le pays pour s’enrichir, a achevé de plomber notre réputation sur place. La France a également hébergé le fils Duvalier, dit Baby Doc, durant vingt cinq ans, alors même qu’il était recherché pour crimes contre l’humanité. Avec un tel passif, autant dire que la population haïtienne n’attend pas grand chose de la France est donc positif que la MMAS, chargée de rétablir la sécurité en Haïti, ait été placée sous le commandement du Kenya. Au travers de cette résolution, nous affirmons notre soutien à cette initiative, nécessaire pour mettre un terme au règne des gangs et permettre la bonne distribution de l’aide humanitaire. Néanmoins, comme nous l’ont rappelé les précédentes missions des Nations unies déployées sur place, nous devrons rester vigilants pour faire en sorte que les forces kenyanes ne commettent pas d’exécutions sommaires, comme le craignent les observateurs.

La capitale est à l’arrêt : écoles et commerces sont fermés, les habitants contraints à l’angoisse ou à l’exil. Des commissariats sont attaqués, des prisons vidées et des familles entières jetées sur les routes. Un an après la mise en place du Conseil présidentiel de transition, les espoirs s’essoufflent et les bandes armées élargissent encore leur emprise. Ce qui se joue aujourd’hui en Haïti n’est pas une crise passagère. C’est une détresse durable, une menace régionale et un appel à la responsabilité internationale. Depuis plusieurs années, nous suivons avec inquiétude la dégradation continue de la situation en Haïti. Mais aujourd’hui, ce n’est plus l’inquiétude qui domine : c’est l’urgence. Le Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, M. Volker Türk, a récemment parlé d’un « nouveau point de crise » pour les droits humains en Haïti. Cette expression lourde de sens résume à elle seule l’ampleur de la catastrophe en cours un État affaibli, des gangs qui prennent le contrôle de territoires entiers, une population prise en étau entre la violence et l’abandon. Au travers de cette proposition de résolution, nous affirmons une position claire : la communauté internationale ne peut plus rester spectatrice. La France, en tant que nation présente dans la Caraïbe, a une responsabilité particulière. Nos territoires ultramarins, Saint Martin au premier chef, sont aux avant postes de cette proximité. Je veux ici redire ma solidarité avec le peuple haïtien, confronté à une crise d’une intensité exceptionnelle. Cette solidarité est d’autant plus forte que, à Saint Martin, nous vivons cette réalité au plus près. La communauté haïtienne y est nombreuse, active, enracinée et profondément inquiète pour ses proches. Notre île, située à quelques encablures d’Haïti, ressent chaque onde de choc de cette crise. Nous partageons des liens humains, familiaux et économiques. Nous ne pouvons être indifférents. de résolution que nous examinons appelle au déploiement effectif de la Mission multinationale d’appui à la sécurité, sous l’égide des Nations unies. Elle souligne la nécessité de renforcer la coopération policière et d’agir contre la prolifération des armes. Elle soutient également le processus politique engagé sous l’égide de la Communauté caribéenne. Ces orientations sont justes. Elles doivent désormais se traduire par des actes, car chaque jour compte. Il est de notre devoir de rester fidèles à nos valeurs, de ne pas détourner le regard et d’agir, avec humanité,

C’est pourquoi personne ne peut regarder ailleurs, alors que le pays s’enfonce dans une crise sécuritaire, alimentaire et économique majeure. Hier, le ministre de l’intérieur Bruno Retailleau a qualifié la situation de chaotique et réaffirmé l’engagement de la France aux côtés d’Haïti. Je salue la présence du chargé d’affaires d’Haïti nos tribunes. La proposition de résolution invitant à favoriser la restauration de la sécurité en Haïti, afin de créer les conditions nécessaires à la mise en place d’un processus politique de sortie de crise, nous offre une nouvelle occasion de réaffirmer

Parler d’Haïti, c’est aussi garder en tête que sa situation actuelle, tout comme son devenir, nous concerne universellement, car c’est elle qui a fait entrer la démocratie et la liberté dans l’universalité. Plus immédiatement, Haïti se situe à 900 kilomètres de la France, soit à la distance qui sépare Paris de Rome. C’est pourquoi, monsieur le ministre, aider Haïti, c’est aider les outre mer. Plus de 150 000 Haïtiens, qui sont parfois français, vivent aussi dans ces territoires. Tout porte à croire que la violence à laquelle les gangs lourdement armés soumettent Port au Prince est alimentée et soutenue par des cartels du narcotrafic. Nous ne saurions donc laisser se créer dans la Caraïbe, si près de nous, un véritable de la drogue et des armes, selon l’image très juste de Pascal Perri. Certes, tort que Haïti est trop souvent résumé à Port au Prince, mais il n’en reste pas moins que, si l’arrière pays n’est pas en proie au même niveau de violence, la situation de la capitale embolise tout le pays. Les considérants de la proposition de résolution identifient les défis principaux qu’affronte Haïti, au delà du défi sécuritaire. Le nombre des personnes déplacées avoisine 1 million, sur les 3 millions que compte Port au Prince. La part des personnes vivant sous le seuil de pauvreté, en situation d’extrême pauvreté, avoisine la moitié de la population, soit 6 millions de personnes. L’élection de Donald Trump a suscité de nombreuses incertitudes qui pourraient se traduire par un retrait de l’aide budgétaire américaine, resserrant un peu plus l’étau des difficultés sur le pays. Il ne faudrait pas que les devises qui viendraient à manquer en Haïti soient remplacées par la liquidité issue des trafics. Surtout, le danger extrême auquel les enfants sont exposés, à lui seul, doit nous obliger, s’il en était besoin, à agir. le rapport d’Amnesty International est accablant et atroce. Il faut rétablir la sécurité en Haïti. Mais, comme le soulignait le professeur Jean Marie Théodat, nous sommes à cet égard devant un choix cornélien. La part des mineurs dans les gangs est évaluée à environ 30 %. Comment, d’un point de vue moral, voire civilisationnel, engager l’armée contre des enfants ? C’est dire la complexité La mission multinationale d’appui à la sécurité, pilotée par le Kenya, n’a pas été en mesure de tenir ses promesses. Nous connaissons l’engagement de la France au sein des instances internationales en faveur du rétablissement de l’ordre en Haïti, mais nous invitons à l’amplifier, de sorte qu’il débouche sur une force internationale de maintien de la paix sur le fondement du chapitre V de la Charte des Nations unies. L’urgence est déclarée. Sans sécurité, le développement du pays ne pourra être engagé. Là aussi, la présente proposition de résolution doit nous inciter à ne pas occulter que le rétablissement de la sécurité ne saurait être le seul horizon. À l’heure des bouleversements internationaux que nous vivons, et alors que la problématique de la souveraineté alimentaire se pose de manière criante, nous devons aussi regarder Haïti comme un territoire d’une grande fertilité agricole et disposant d’une jeunesse à laquelle il faut redonner espoir.

entre Haïti et la France. Ce moment nous oblige aussi. Privée de l’équivalent de trois années de revenu national, la jeune République, en 1825, n’a pas pu consacrer ses ressources à la construction d’institutions assez solides pour résister aux contingences de l’histoire.

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, il est important pour moi d’être aujourd’hui face à vous pour redire avec force le soutien de la France au peuple haïtien, qui traverse l’épreuve de la violence et du chaos imposés par une véritable guerre des gangs. La France est un État caribéen, comptant des territoires voisins d’Haïti. Nous sommes donc solidaires des défis sécuritaires que ce pays affronte et qui ont des répercussions à l’échelle de toute la région. C’est pourquoi je remercie la sénatrice Hélène Conway Mouret de son engagement sur ce sujet si important. Je tiens aussi à saluer l’engagement continu du groupe d’amitié France Caraïbes en faveur d’Haïti, dont témoigne cette proposition de résolution. Je veux également saluer l’engagement et le sang froid de notre ambassadeur à Port au Prince et de toute son équipe diplomatique ; j’y reviendrai. Après l’assassinat du président Jovenel Moïse, en juillet 2021, et l’éviction du Premier ministre Ariel Henry, en mars 2024, Haïti est désormais entré dans une phase de transition politique. Cela s’est matérialisé par l’accord du 3 avril 2024 et la mise en place d’un exécutif bicéphale, composé d’un conseil présidentiel de transition et d’un gouvernement. Ce dernier a deux priorités : libérer la population de l’emprise des gangs et organiser des élections générales. Je rappelle que le pays n’en a pas connu depuis 2016. La France soutient les autorités de transition haïtiennes et leur agenda. C’est pourquoi, en 2024, nous avons versé 750 000 euros à l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) pour accompagner le processus électoral. Seul le bon déroulement des élections pourra donner une légitimité suffisante au futur gouvernement haïtien. Pour l’heure, la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader. La coalition de gangs a plongé le pays dans un terrible cycle de violence : plus de 5 600 morts et 1 million de déplacés rien qu’en 2024, auxquels s’ajoutent déjà 1 000 morts et 78 000 déplacés depuis le début de l’année 2025. Le 1 avril, avec l’assaut contre la prison de Mirebalais, qui a causé l’évasion de 500 détenus, la violence a franchi un nouveau seuil. Au delà de Port au Prince et du département de l’Artibonite, c’est désormais l’ensemble du territoire national qui est menacé. nationales de sécurité, constituées de 10 000 hommes et bénéficiant du soutien d’une force multinationale, ne parviennent pas à contenir cette violence. Cette insécurité empêche l’acheminement de l’aide humanitaire et prive les Haïtiens de l’accès aux services de base : santé, éducation, alimentation. Aujourd’hui, 5,5 millions d’Haïtiens, soit la moitié de la population, souffrent de la faim. Face à cette urgence, la France est pleinement engagée. Elle est, avec l’Espagne, le seul État membre de l’Union européenne encore présent à Port au Prince. En 2024, l’aide française a représenté 40 millions d’euros de dons, faisant de nous le troisième bailleur d’Haïti, derrière les États Unis et le Canada. Des liens indéfectibles unissent nos deux pays. Nous avons en partage une histoire, une géographie et une langue. Nos relations diplomatiques sont étroites le 29 janvier dernier, le Président de la République a reçu à Paris le président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire ; je me suis pour ma part entretenu avec mon homologue, Jean Victor Harvel Jean Baptiste. Notre priorité, c’est le rétablissement de la sécurité. Depuis 2023, nous avons mobilisé plus de 11 millions d’euros pour soutenir la mission multinationale d’appui à la sécurité, la police nationale et les forces armées haïtiennes. Cet appui devra s’accompagner d’une montée en puissance des forces de sécurité et d’une lutte plus ferme contre les trafics et la corruption. À ce stade, le Secrétaire général des Nations unies a écarté l’option, sollicitée par en opération de maintien de la paix, pour privilégier le renforcement de la MMAS sur le modèle somalien. La France est favorable à une plus grande implication des Nations unies et nous nous tenons prêts à agir en ce sens au Conseil de sécurité. Nous agissons pour la mise en place de sanctions à l’encontre des chefs de gangs et de ceux qui les financent. À l’ONU, la France a soutenu l’adoption d’un régime de sanctions spécifiques. Nous sommes à l’origine des sanctions mises en place par l’Union européenne en juillet 2023. Trois chefs de gangs ont déjà été désignés en décembre 2024 et de nouveaux dossiers préparés par mes équipes sont en cours d’examen Sur le plan humanitaire, la France a alloué à Haïti 16,5 millions d’euros d’aide en 2024. Quelque 8,5 millions d’euros ont été consacrés à l’aide alimentaire, essentiellement les cantines scolaires, avec une politique de soutien aux producteurs haïtiens. pour les migrations), d’aider les migrants haïtiens expulsés de République dominicaine. Plus de 16 millions d’euros ont été consacrés à des projets de développement développement (AFD) et Expertise France, notamment dans les domaines de la santé maternelle et infantile, de l’éducation et de l’agriculture. Un million d’euros ont également été alloués à notre coopération culturelle et éducative. Aujourd’hui, plus de 4 000 étudiants haïtiens poursuivent leurs études dans des établissements de l’Hexagone, mais aussi en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane.

À l’occasion de son entretien avec Leslie Voltaire, le 29 janvier dernier à l’Élysée, le Président de la République a indiqué que notre passé commun ne devait pas être oublié et qu’il était de la responsabilité de la France de faire vivre la mémoire de l’esclavage sur l’ensemble du territoire national, comme en Haïti. Des initiatives seront annoncées par le Président de la République le 17 avril prochain, date éminemment symbolique, puisque c’est par l’ordonnance de Charles X du 17 avril 1825 que la France a concédé la reconnaissance de l’indépendance d’Haïti, en contrepartie d’une indemnité. À ce sujet, je le dis très clairement, la France est ouverte à un dialogue apaisé sur les questions mémorielles. Enfin, nous ne pouvons ignorer la décision de l’administration américaine de geler son aide internationale. représentait 60 % de l’aide humanitaire reçue par Haïti. À cela s’ajoute le fait que les expulsions d’Haïtiens en situation illégale depuis les États Unis ont commencé. Pour notre part, en dépit des restrictions budgétaires, nous avons la ferme intention de continuer à soutenir Haïti et sa population en 2025. Je voudrais, avant de conclure, avoir un mot pour nos presque 1 000 compatriotes présents sur place, qui craignent pour leur sécurité et dont les enfants poursuivent péniblement leur scolarité sur Zoom. tiens également à rendre un hommage appuyé à notre ambassadeur et à nos agents sur place, qui travaillent dans des conditions extrêmement dégradées : célibat géographique imposé déplacement dans des véhicules blindés précédés par des drones de reconnaissance ; évacuation des bureaux de l’ambassade qui se trouvaient à portée des échanges de tirs entre les gangs et la police.

Plus que jamais, les Haïtiennes et les Haïtiens ont besoin du soutien de la France pour obtenir le retour à la stabilité. Je resterai pleinement engagé sur ce sujet et je sais pouvoir compter sur votre mobilisation. La discussion

proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République national anticriminalité organisée, sont chacune parvenues à l’adoption d’un texte commun.

et à la souveraineté audiovisuelle, et, en conséquence, le retrait de la suite de la proposition de loi sur la profession d’infirmier inscrite le mardi 6 mai ; l’inscription en premier point de l’ordre du jour du mardi 6 mai d’une déclaration suivie d’un débat, en application de l’article 50 1 de la Constitution, portant sur la souveraineté énergétique de la France ; l’inscription en deuxième point de l’ordre du jour du mardi 6 mai de la deuxième lecture de la proposition de loi portant reconnaissance par la Nation et réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982, et, en conséquence, le retrait de la suite de cette deuxième lecture inscrite le mercredi 7 mai l’inscription en deuxième point de l’ordre du jour du mercredi 7 mai de la suite éventuelle de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé.

pour un sénateur non inscrit. Le délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat pourrait être fixé au lundi 5 mai à quinze heures. Il n’y a pas d’opposition ?… Il en est ainsi décidé.

des politiques françaises et européennes de régulation des plateformes en ligne ? » Je vous rappelle que, dans ce débat, le Gouvernement aura la faculté, s’il le juge nécessaire, de prendre la parole immédiatement après chaque orateur pour une durée de deux minutes l’orateur disposera alors à son tour du droit de répartie, pour une minute. Madame la ministre déléguée, vous pourrez donc, si vous le souhaitez, répondre après chaque orateur, une fois que celui ci aura retrouvé une place dans l’hémicycle.

nos choix politiques ou, au contraire, notre apathie peut tous nous emporter dans une grande bascule ou provoquer le sursaut qui protégera nos démocraties. Oui, nos démocraties libérales, telles qu’elles se sont développées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, sont aujourd’hui menacées par la montée des régimes autoritaires, illibéraux ou impérialistes qui, piétinant le droit international et le multilatéralisme, voient dans nos systèmes une entrave à leur expansion et un contre modèle qui leur est insupportable. Leur travail de sape passe aujourd’hui par la promotion de tout ce qui fracture nos sociétés et par la manipulation du débat public. rien de nouveau. Tout tenait déjà dans le fameux paradoxe de la tolérance de Karl Popper : « La tolérance illimitée ne peut que conduire à la disparition de la tolérance. […] Si nous ne sommes pas prêts à défendre une société tolérante contre les assauts des intolérants, alors les tolérants seront détruits, et la tolérance avec eux. » Pour mener leur offensive, les adversaires de la démocratie se

La déstabilisation du débat public a progressé, par ce biais, à une échelle industrielle. En effet, ces plateformes numériques sont devenues les nouvelles infrastructures de notre quotidien. Elles ne sont plus de simples services, mais les espaces les espaces incontournables de nos relations sociales, de notre accès à l’information, de nos loisirs, de nos achats et même de nos opinions. Aujourd’hui, des milliards de personnes dans le monde dépendent de Google pour chercher, de YouTube pour comprendre, de Facebook pour échanger, de TikTok de X pour s’informer – ou se désinformer. Au travers de ces plateformes, ceux que Giuliano da Empoli appelle les « ingénieurs du chaos », ces idéologues au service des dirigeants autoritaires, accumulent des données et abusent des algorithmes pour diviser profondément

Nous devons porter un regard critique sur ce capitalisme de la donnée ou ce « capitalisme de surveillance », pour reprendre les termes de Shoshana Zuboff. Les plateformes orientent le débat public en fonction de leurs propres intérêts économiques ou idéologiques. Ce que nous voyons sur nos écrans n’est pas un reflet neutre de l’opinion, mais un résultat rangé, ordonné et optimisé de la captation de nos données : optimisé pour garder notre attention, pour nous faire « scroller » à l’infini, « liker » et consommer. Les plateformes sont devenues des éditeurs sans le dire. Elles filtrent, classent, favorisent certains contenus et en invisibilisent d’autres, selon des logiques que personne ne peut vraiment voir, donc contester. Et ce n’est plus gratuit ! Nous payons avec ce que nous avons de plus intime : nos données, nos comportements et notre attention. Le marché mondial de la publicité numérique pèse plus de 600 milliards de dollars par an. Mais au delà de cette marchandisation de l’intime, c’est notre démocratie elle même qui est désormais fragilisée. L’ingérence des plateformes dans le débat public prend deux formes principales. La première, la plus visible, est celle de la désinformation.

qui impose des obligations strictes aux très grandes plateformes, et que nous avons nous mêmes transposé dans la loi pour sécuriser et réguler l’espace numérique. Nous disposons donc d’un panel d’outils que je pense pour partie robustes. L’heure est venue de les mettre en œuvre. La loi ne vaut que si elle est appliquée avec rigueur. Il faut mettre fin à l’impunité numérique. La seconde forme d’ingérence, plus insidieuse, plus difficile à détecter, est celle des algorithmes. Chaque plateforme décide, au travers de ses propres formules couvertes par le secret industriel, de ce que vous allez voir ou non. Ce n’est pas anodin compte tenu de la place qu’elles ont prise dans nos vies : c’est un façonnage du réel. Les algorithmes créent des bulles, des chambres d’écho, structurent l’opinion, orientent à partir des émotions, polarisent le débat. Et dans certains cas, ils sont délibérément utilisés pour influencer des processus électoraux, affaiblir des sociétés, déstabiliser des régimes, comme cela a été le cas en Moldavie, en Géorgie ou dans les Balkans, où les manipulations

se fait pas pour autant dans l’ombre. Le rachat de X par Elon Musk et sa mise à la disposition de la machine électorale de Trump, ainsi que son soutien aux partis d’extrême droite européens, se font au su et au vu de tous. On connaissait la manipulation des algorithmes due à des ingérences extérieures ; désormais, c’est le dirigeant de la société lui même qui manipule sa plateforme, mettant un terme à toute forme de modération et, par la même occasion, mettant fin à l’illusion de la neutralité. Avec le retour de cette rhétorique toxique, toute régulation est vue comme une atteinte à la liberté d’expression. Comme si modérer les plateformes revenait à museler le peuple ! C’est un contresens dangereux. Car réguler ne revient pas, comme le disent les trumpistes, à manipuler l’opinion ou à faire taire qui qui que ce soit. Au contraire, et grâce à des règles communes, c’est préserver l’essence même de la démocratie, à savoir le débat libre et éclairé, dans sa diversité, sa pluralité et la possibilité de délibérer sans être manipulé par les grandes entreprises ou le mensonge. Dans ce contexte, notre large dépendance aux outils, services et infrastructures numériques, notamment américains, doit être remise en cause. Alors, que faire ? Sur la désinformation, le cap est clair : la France doit pousser l’Europe à appliquer de manière stricte, rapide et implacable le DSA, dès que les faits sont avérés. bec et ongles notre souveraineté numérique. Chaque violation doit être sanctionnée et chaque manquement exposé publiquement. Sur les algorithmes, il reste beaucoup à faire. Le DSA prévoit quelques outils. Pour lutter contre l’effet « boîte noire » des algorithmes, nous devons encourager les audits indépendants autorisés par le DSA. Nous aimerions vous entendre à ce sujet, madame la ministre déléguée. Nous avons besoin d’une expertise publique, scientifique et indépendante, pour comprendre et contrôler ces outils qui structurent notre vie collective nous prémunir en urgence des ingérences, tout en garantissant un espace démocratique d’expression. La tâche est ardue : elle appelle à faire d’abord preuve de lucidité, puis de détermination. Ce combat pour défendre le débat public n’est pas secondaire. Il est central et urgent : c’est la raison pour laquelle nous ouvrons le débat aujourd’hui.

Madame la présidente, madame la ministre déléguée, mes chers collègues, je vous remercie sincèrement de cette discussion sur la sincérité du débat public et la régulation des plateformes.

Que penser aussi de ce qui est arrivé à Arthur, 22 ans, qui s’est pendu après un changement de genre intervenu à l’âge de 16 ans, perturbé par une prétendue idéologie de liberté ? Elle s’appelait Célia, et ses parents ont clairement pointé la responsabilité des réseaux sociaux tant dans sa volonté de changer de genre que dans sa volonté

C’est à nous, législateurs, d’être fermes et de ne pas faiblir devant ces concepts de pseudo liberté et de pseudo libre expression. Personnellement je considère que nous et nos enfants sommes attaqués par des groupuscules de fanatiques. C’est aussi valable pour notre économie : mensonges et sont véhiculés par des marchands de peur qui s’en prennent à toutes les strates de nos institutions et à nos valeurs. et à nos valeurs. À l’échelle de l’Union européenne, l’arsenal normatif concernant les plateformes s’est étoffé au cours des dernières années. Afin de limiter la propagation des, l’adoption du DSA a marqué un véritable tournant dans la législation européenne. Il oblige les très grandes plateformes à faire la lumière sur leurs systèmes de recommandation de contenus auprès de leurs utilisateurs. Les plateformes ont ainsi pour obligation d’évaluer et de prendre des mesures pour atténuer les risques qui découlent de l’utilisation de leurs services. La Commission européenne a également demandé à huit des principales plateformes de fournir des explications sur la prolifération de vidéos trompeuses par lesquelles on peut attribuer à un individu des comportements qui ne sont pas les siens grâce à l’intelligence artificielle. En effet, les réseaux sociaux ne peuvent être considérés comme une simple courroie de transmission. Nous devons tous avoir un leitmotiv responsabiliser et contraindre les plateformes et les empêcher, avec des outils justes et équilibrés, de se soustraire, de quelque manière que ce soit, à leurs obligations. leurs obligations. Certes, nous en avons tous conscience, cet exercice est particulièrement complexe, tant nous devons répondre simultanément à deux exigences de taille : l’identité numérique pour protéger nos enfants ; la garantie d’une véritable traçabilité et la véracité des informations diffusées par les plateformes.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens à mon tour à remercier nos collègues écologistes d’avoir inscrit à l’ordre du jour de nos travaux sujet qui pose certainement beaucoup plus de questions qu’il n’apporte de réponses. Le réseau internet et le développement des plateformes numériques ont eu des bienfaits considérables sur notre société, notamment en renforçant le lien social et l’accès aux connaissances. Cependant, comme la plupart des grandes innovations technologiques, le numérique est porteur de progrès, mais également facteur de dangers. Nous vivons en effet à une époque où la communication est plus accessible que jamais, mais où la désinformation et la manipulation de l’information menacent la sincérité du débat public. La régulation des plateformes en ligne, au niveau tant français qu’européen, est essentielle pour garantir la qualité des échanges démocratiques. Je vais tenter d’exposer les politiques mises en œuvre et les défis à relever pour promouvoir un environnement numérique sain. Les plateformes en ligne, telles que les réseaux sociaux et les moteurs de recherche, jouent un rôle central dans la diffusion de l’information. Elles peuvent favoriser la participation citoyenne, mais elles sont également le vecteur de fausses informations et de discours de haine. Les données montrent que les contenus manipulés ont souvent plus de visibilité que ceux qui respectent les faits. Ce constat appelle une action rapide et coordonnée. Les réseaux sociaux sont devenus des espaces de désinformation, de manipulation et d’ingérence, en offrant un cadre favorable à la propagation de fausses nouvelles. Par parenthèse, se pose aussi la question de l’anonymat sur ces plateformes. J’aurai l’occasion, madame la ministre, de formuler quelques propositions en la matière dans quelques semaines. Il me paraît en effet urgent d’apporter des solutions, afin de protéger les utilisateurs et de leur permettre d’utiliser des outils sécurisés et fiables. On ne peut accepter plus longtemps de vivre dans une zone où la protection diffère du monde réel. De surcroît, internet et les réseaux sociaux constituent la principale source d’information pour un Français sur deux. La désinformation a pris de l’ampleur pendant le confinement et la crise sanitaire, au cours desquels les réseaux sociaux se sont fait la caisse de résonance de théories complotistes. Les groupuscules extrêmes trouvent dans cet outil de communication un nouveau moyen de diffuser leurs idées, y compris pour déstabiliser la démocratie représentative. On a pu mesurer, en Europe et aux États Unis, le risque majeur que font peser les réseaux sociaux sur les processus électoraux. Lors des dernières élections américaines, le nombre de faits inexacts qui ont été propagés a progressé à un niveau jusqu’alors jamais atteint. Une étude de la revue en 2018 montre que les fausses informations,

a 70 % de chances de plus d’être reprise qu’une information vraie. Ces dérives sont facilitées par le mode de fonctionnement des plateformes. En effet, leur modèle économique repose sur des recettes publicitaires proportionnelles au trafic suscité par les utilisateurs. Pour accroître le temps de présence des utilisateurs et multiplier les gains publicitaires, les algorithmes des plateformes mettent en avant les contenus les plus virulents et les moins nuancés.

Dans un tel contexte, est il encore possible de garantir la sincérité du débat public ? En France, la loi de 1881 a fixé un cadre législatif pour l’exercice de la liberté d’expression,

il est crucial de garantir que ces régulations ne portent pas atteinte à la liberté d’expression. De plus, la réponse ne pouvait rester nationale face à des géants du numérique à la capacité d’influence planétaire. Le législateur européen est intervenu en adoptant le règlement sur les services numériques (DSA), applicable depuis le 17 février 2024. ci vise une responsabilisation des plateformes. Il prévoit en particulier de nombreuses mesures graduées selon les acteurs en ligne, en fonction de la nature de leurs services et de leur taille. Les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche sont soumis à des exigences plus strictes. Lorsqu’un signalement est effectué, ils doivent rapidement retirer ou bloquer l’accès au contenu illégal. Dans ce cadre, ils coopèrent avec des « signaleurs de confiance » présents dans chaque pays. En outre, les plateformes doivent rendre plus transparentes leurs décisions en matière de modération des contenus et proposer un système de recommandation de contenus non fondés sur le profilage. En France, le coordinateur national est l’Arcom, comme l’a prévu la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique. En cas de non respect du DSA, des astreintes et des sanctions peuvent être prononcées. Pour les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche, la Commission européenne peut infliger des amendes allant jusqu’à 6 % de leur chiffre d’affaires mondial. En cas de violations graves et répétées, les plateformes peuvent même se voir interdire leurs activités sur leur marché européen. Néanmoins, quelle efficacité ont ces mesures ? Depuis l’adoption du DSA, seize enquêtes ont été diligentées par la Commission européenne à l’encontre des très grandes plateformes en ligne. Jusqu’à présent, une seule, pour manquement à l’encontre de TikTok, a permis le retrait de l’un des programmes Le 18 décembre 2023, la Commission européenne a également ouvert une procédure formelle d’infraction à l’encontre du réseau social X pour manquement aux règles européennes. En juillet 2024, elle a estimé dans les conclusions préliminaires de cette enquête que X enfreignait ses obligations en matière de modération des contenus illégaux et de lutte contre la désinformation, en particulier les obligations de transparence concernant les publicités diffusées et l’accès des chercheurs aux données de la plateforme. Enfin, en Enfin, en juillet 2025, la Commission européenne a annoncé des mesures techniques supplémentaires auprès de la plateforme. Pour le moment, les pouvoirs d’enquête et de contrôle dont dispose la Commission européenne semblent insuffisamment utilisés. La procédure doit suivre un long cheminement avant que toute non conformité ne soit prononcée. Aussi est ce avec la plus grande attention que nous écouterons vos conclusions et propositions sur le sujet, madame la ministre. L’efficacité de la mise en œuvre du règlement européen reposera sur un partage efficace d’informations, d’expériences et de compétences entre la Commission et les autorités nationales, lesquelles devront elles mêmes être dotées de moyens suffisants. Plusieurs défis restent à relever. Tout d’abord, l’application effective de ces régulations sera cruciale. Les plateformes doivent être tenues responsables de leurs actions, mais cela nécessite des ressources et implique une coopération étroite entre États membres. Ensuite, la question de la transparence et de l’impartialité des algorithmes reste centrale. Comment garantir que ces systèmes ne favorisent pas certaines voix au détriment d’autres ? Pour conclure, la sincérité du débat public dépend étroitement de nos actions collectives en matière de régulation des plateformes en ligne. Les politiques adoptées, qu’elles soient françaises ou européennes, doivent être rigoureusement appliquées et constamment adaptées aux évolutions technologiques.

la sincérité du débat public à l’ère numérique et la manière dont les politiques françaises et européennes régulent les plateformes en ligne pour garantir un espace d’échange authentique et respectueux des valeurs démocratiques. Les plateformes numériques ont acquis une place centrale dans notre vie sociale, politique et économique. Elles constituent un espace d’échange et de débat, mais également un terrain de manipulation, où les frontières entre la réalité et le mensonge sont souvent floues. Le phénomène de la désinformation a pris une ampleur considérable. Au delà des simples erreurs d’information, des campagnes de manipulation sont systématiquement menées pour influencer les opinions publiques, perturber les processus électoraux et déstabiliser des sociétés entières.

en donnant une image positive de l’invasion russe en Ukraine. Je pourrais également citer les multiples campagnes de désinformation autour du covid 19, de l’élection présidentielle américaine ou des élections européennes. La désinformation est grave pour notre démocratie.

Les plateformes numériques sont devenues les vecteurs privilégiés de la diffusion de discours haineux, de propos diffamatoires ou de pratiques de harcèlement. L’un des fondements de ces abus réside dans l’anonymat

comme une garantie de la liberté d’expression, il peut également servir de bouclier à ceux qui souhaitent propager la haine, la violence et la désinformation. Les avis sur cette question sont divers.

En offrant un refuge aux comportements nuisibles, l’anonymat permet à des individus de diffuser des informations fausses ou des propos haineux sans craindre des représailles. Il est donc crucial de poser la question d’une éventuelle identification des utilisateurs sur les plateformes en ligne pour prendre à bras le corps le problème de l’impunité sur internet. D’un côté, l’obligation de dévoiler son identité en ligne permettrait à nos forces de l’ordre et à la justice d’agir plus efficacement

Au delà de la question de l’anonymat, nous devons évidemment poursuivre nos efforts pour réguler les plateformes numériques dans leur globalité. Comme l’ont rappelé les orateurs précédents, l’Union européenne a déjà entrepris

visent à renforcer la transparence, à protéger les utilisateurs et à prévenir les abus des géants du numérique. Le DSA impose aux plateformes une série d’obligations en matière de modération des contenus, de transparence des algorithmes et de coopération avec les autorités de régulation, pour lutter contre les contenus illégaux. Le DMA renforce la compétitivité des marchés numériques, en luttant contre les pratiques anticoncurrentielles des géants du secteur.

La France et l’Union européenne doivent donc veiller à ce que leurs efforts de régulation aboutissent à un mécanisme de responsabilité protégeant davantage les utilisateurs contre les abus et garantissant un espace numérique plus sûr et plus transparent.

je remercie mes collègues du groupe GEST d’avoir proposé ce débat. Il est essentiel que nous éclaircissions cette question éminemment politique : comment garantir, à l’ère numérique, la liberté et la sincérité du débat public ? Plus encore, comment faire en sorte que les plateformes respectent les principes fondamentaux de notre modèle républicain et démocratique ? Les plateformes numériques – réseaux sociaux, moteurs de recherche, agrégateurs de contenus – occupent une place prépondérante dans nos vies.

faire face, notre arsenal législatif est insuffisant. La commission d’enquête conduite par nos collègues Dominique de Legge et Rachid Temal l’a clairement établi, la France est aujourd’hui vulnérable face aux ingérences numériques étrangères. Leur rapport souligne une absence de stratégie coordonnée et pointe les failles de notre système de réponse. Aussi proposent ils une évolution ambitieuse : reconnaître le rôle actif des grandes plateformes en les requalifiant comme des acteurs éditoriaux responsables. Cette requalification aurait une portée juridique majeure

Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk et sous couvert d’une liberté d’expression sans filtre, des comptes pourtant sanctionnés pour incitation à la haine ont été réintégrés. Les plateformes sont néfastes pour les mineurs lorsqu’elles les exposent à des contenus anxiogènes, sexualisés ou promouvant des comportements dangereux. Pire encore, les algorithmes de recommandation les enferment dans des boucles de contenus addictifs et délétères pour leur santé mentale. Nous le savons, l’efficacité des mécanismes de modération actuels reste très insuffisante. Le rapport annuel pour 2023 de l’Arcom l’avait bien les pratiques de retrait des contenus haineux sont incohérentes. L’opinion publique ne doit pas être structurée par des systèmes automatisés, sans transparence ni contrôle démocratique. Mes chers collègues, la libre formation de l’opinion nécessite un socle commun de vérité. Il est urgent que nous nous saisissions des propositions issues de la commission d’enquête, pour définir une doctrine nationale de lutte contre les manipulations de l’information et pour articuler efficacement la coopération entre les services de renseignement et les autorités de régulation. Les plateformes numériques ne peuvent plus être considérées comme de simples hébergeurs techniques. À cet égard, le DSA, adopté le 19 octobre 2022, marque une avancée importante. a introduit des obligations de transparence sur les algorithmes, des exigences de retrait rapide des contenus manifestement illicites, ainsi qu’un devoir d’évaluation des risques systémiques pesant sur les très grandes plateformes. Dès lors qu’un système de recommandation favorise les contenus les plus polarisants, il faut le sanctionner, sans pour autant céder à des réflexes d’urgence et de facilité. internet, dite loi Avia, dont la disposition phare a été censurée par le Conseil constitutionnel en 2020. Nous devons obtenir un droit d’accès réel aux mécanismes de construction de ces algorithmes. C’est une condition essentielle pour comprendre les dynamiques de diffusion et redonner du sens à la régulation. Enfin, nous avons besoin d’une autorité de régulation disposant de moyens réels, capable de formuler des recommandations contraignantes et de faire respecter la loi.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l’arrivée d’internet, puis, dans les années

la Chine et maintenant les États Unis. Les propriétaires des plateformes ne se gênent pas pour modifier leur algorithme et faire ouvertement campagne pour des candidats d’extrême droite. Ne soyons pas naïfs, les élites de la tech ont bien un projet politique

L’intelligence artificielle amplifie encore les menaces. Les hypertrucages prolifèrent et sèment la confusion. Demain, les se substitueront aux moteurs de recherche et aux plateformes et choisiront les vérités qu’elles voudront bien

la DG Connect, doit utiliser la faculté qui lui est offerte de procéder à des inspections dans les locaux des plateformes. De même, les chercheurs indépendants doivent réellement pouvoir accéder aux données des très grandes plateformes, qui restent des boîtes noires.

des risques associés au développement non régulé de l’IA pour l’information fiable, de la prolifération de faux sites d’information automatisés, ou encore de la désinformation infiltrée dans les. En outre, la question des droits fondamentaux et celle des risques systémiques pesant sur l’intégrité des élections démocratiques

Ce média incarne pourtant la première ligne de défense informationnelle dans des pays frontaliers de l’Union européenne, tels que la Géorgie et l’Azerbaïdjan. Madame la ministre,

dans le respect du pluralisme et la confrontation des idées. Nous le savons tous, l’intégralité des productions de la presse a été pillée sans vergogne par les plateformes de l’intelligence artificielle,

– pillent ces ressources avec la même rapacité qui pousse Donald Trump à vouloir s’emparer des terres rares ukrainiennes. Nous sommes entrés dans l’économie de la rapine. Les Gafam ont porté au pouvoir l’actuel président des États Unis. Ils entendent maintenant engranger les dividendes de leur investissement. Ils souhaitent abolir toute règle susceptible d’entraver le pillage méthodique et inextinguible des ressources de l’esprit. Dans un mémorandum adressé à la Maison Blanche le 13 mars dernier, les dirigeants d’OpenAI demandaient à l’administration américaine de tout mettre en œuvre pour en finir avec la propriété intellectuelle en Europe, tout particulièrement ici, en France.

les États Unis dégagent un excédent de 137 milliards d’euros dans le domaine des services, notamment dans celui du numérique, où l’Europe est très faible.

comme l’explique si justement Maria Ressa, prix Nobel de la paix, « si on laisse les mensonges se propager plus vite que les faits, notre réalité sera divisée, la réalité partagée sera brisée, et le journalisme et la démocratie deviendront impossibles

Nous devons notamment exiger une modération humaine et journalistique des contenus, une transparence accrue des algorithmes et l’encadrement strict de l’utilisation des . La régulation des plateformes existantes doit être la première jambe de notre action collective, la seconde consistant à favoriser la création de nouvelles plateformes numériques européennes.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l’avènement d’internet portait en lui une promesse d’émancipation par la connaissance, d’ouverture au dialogue universel et d’éclosion d’une intelligence collective. Or cette vision s’est progressivement obscurcie, cédant la place à l’enfermement dans un espace numérique pourtant présenté comme illimité. Au cœur de cette transformation se trouvent les plateformes en ligne, dont le modèle économique, fondé sur la captation de l’attention, tend à maximiser le temps qu’y passent les utilisateurs. Cette course incessante à l’attention, dictée par une logique marchande, favorise la diffusion de contenus sensationnalistes, polémiques, voire fallacieux. Parallèlement, les algorithmes de recommandation, loin de favoriser une information équilibrée, exacerbent la propagation des fausses nouvelles à une échelle inédite. Ils accentuent la polarisation du débat public en enfermant les utilisateurs dans des bulles de filtre. Ce modèle a conféré aux plateformes un pouvoir de manipulation lui même inédit, non seulement en raison de leur capacité à capter des données personnelles, mais aussi et surtout du fait de leurs algorithmes, qui deviennent de véritables leviers de contrôle. Ces mécanismes servent à la fois les intérêts commerciaux de diverses entreprises et certaines ambitions étatiques, notamment par le biais des législations extraterritoriales.

contre les géants du numérique ? Toutefois, l’application stricte du cadre juridique existant ne suffira pas. Pour garantir la sincérité du débat public face

Il est tout aussi urgent de réformer le régime de responsabilité des plateformes. Celles dont les algorithmes modèlent l’accès à l’information doivent faire l’objet d’obligations comparables à celles que devons garantir la portabilité et l’interopérabilité des données entre plateformes. Il doit s’agir d’un droit effectif, au service des utilisateurs.

des données, s’érigent en nouveaux seigneurs numériques, captant la richesse produite par le travail gratuit des utilisateurs. Madame la ministre, pour rompre avec cette dynamique et renforcer la régulation des plateformes aux échelles nationale et européenne, quelles initiatives

Face aux géants extra européens, il ne suffit pas de poser des garde fous. Il faut être capable d’innover et de produire, ce qui suppose de maîtriser les technologies stratégiques.

Cet effort doit se traduire par un investissement massif dans les infrastructures numériques clés : le quantique, l’, les semi conducteurs, l’informatique en nuage ou encore les supercalculateurs. Un tel travail suppose aussi un changement d’échelle.

technologies et la préférence européenne ? Estimez vous que la France et l’Europe doivent se fixer pour objectif d’accompagner l’émergence de véritables plateformes numériques européennes

de notre époque, celui de la sincérité du débat public dans un espace numérique devenu très souvent, trop souvent, et pour beaucoup de nos concitoyens, le premier lieu d’information et parfois de désinformation, de manipulation, voire d’addiction.

Je sais les formidables chances que représente le numérique dans de nombreux domaines : les avancées scientifiques, l’émancipation et tous les nouveaux usages que le numérique a pu nous apporter au cours des dernières décennies.

donc la réalité en face. La question des plateformes numériques est partie prenante de cette réalité. Elle façonne de plus en plus l’opinion publique et fait la part belle à des contenus parfois trompeurs, que certaines puissances étrangères instrumentalisent pour influencer nos débats ou nos choix, –, dans certains pays de l’Union européenne, nos élections. Les algorithmes jouent un rôle clé dans ces entreprises de désinformation et de manipulation. La santé de notre démocratie ne doit pas dépendre des systèmes de recommandation, qui favorisent les contenus polarisants, outranciers et qui cherchent à capter notre attention en faisant appel à nos émotions les plus négatives. En somme, la recherche de viralité

de la prise de conscience, que je crois collective, des mécanismes de l’attention souterrains et des algorithmes qui ébranlent parfois les piliers de notre société.

de nouveaux pouvoirs d’injonction pour lutter, par exemple, contre les contenus diffusés par des médias qui seraient visés par des sanctions internationales. Je pense enfin au développement de l’éducation aux médias et à l’information,

Oui, c’est le rôle de la France que d’en être le fer de lance, face à des pays, adversaires ou anciens alliés, dont l’objectif est de faire la guerre à nos sociétés multiculturelles, à nos valeurs démocratiques et à nos libertés publiques. Toutefois, la France doit aussi se prémunir d’une forme de dérive. en effet se mettre en place à bas bruit une société d’algorithmes, où des décisions lourdes de conséquences – qu’il s’agisse d’allocations, de contrôles ou de sanctions – sont prises sans transparence, sans recours et sans humanité. Dans nos services publics, des algorithmes sont déjà utilisés pour détecter les fraudes, traquer les chômeurs, hiérarchiser les urgences, le tout dans une logique comptable, punitive et parfois déshumanisée. Par exemple, quelque dix associations, dont

solution, politique, passe par un écosystème numérique européen plus proche de nos valeurs communes. Mon collègue Guillaume Gontard en a esquissé les contours. Je le disais en introduction de ce débat : nous sommes face à un risque de grande bascule. nos démocraties n’en sont pas moins résilientes. Nous devons renforcer leur robustesse, non pas en nous emparant des armes de nos ennemis, mais en faisant la lumière sur les ingérences et les manipulations, ainsi qu’en garantissant la transparence et la modération. du chercheur Hugo Micheron, qui estime que, dans un monde où les attributs de la puissance sont redistribués par la nouvelle donne technologique, il est temps que, aux ingénieurs du chaos, l’Europe puisse opposer les ingénieurs de la démocratie. Très bien